jours, la communauté internationale, y compris la France, se félicite de l’annonce d’un futur traité de paix. Si nous pouvons nous réjouir des efforts réalisés pour installer une paix juste et durable dans la région, nous ne savons à ce stade que très peu de choses sur le contenu de cet accord. nous imaginons que l’Arménie a dû faire de nombreuses concessions. Quoi qu’il en soit, les prisonniers de guerre arméniens retenus à Bakou ne sauraient être les oubliés de ces négociations, comme il semble que ce soit le cas. trois prisonnières et prisonniers arméniens du Haut Karabakh à croupir dans les geôles azerbaïdjanaises. Parmi eux figurent d’anciens dirigeants de l’Artsakh, des journalistes, des militants des droits humains,

une attention toute particulière aux inquiétudes exprimées par les organisations de défense des droits de l’homme quant à l’équité du jugement et au traitement des accusés. Nous avons rappelé à plusieurs reprises – et nous continuerons de le faire

touchent toutefois à la question bien plus vaste de l’instauration d’une paix durable entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. À cet égard, la France a salué l’annonce de l’aboutissement de la négociation d’un traité de paix entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. Plus rien ne s’opposant désormais à sa signature, nous avons appelé les parties à fixer une date sans délai. La normalisation des relations entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, dans le respect de l’intégrité territoriale et de la souveraineté des deux États, doit permettre au Sud Caucase de devenir un espace de paix, d’intégration et de coopération, avec des frontières ouvertes, au bénéfice des populations de la région.

ne s’agit pas simplement d’un conflit de plus dans une région instable ; il s’agit d’une guerre hybride, alimentée par des intérêts économiques, miniers et stratégiques, qui échappe aux logiques classiques des affrontements étatiques ou civils. Il me faut rappeler que le Mouvement du 23 mars (M23), soutenu de manière attestée par le Rwanda, n’est pas un acteur isolé. Il s’inscrit dans une toile complexe d’ingérences, de prédation des ressources naturelles et de reconfigurations d’alliances régionales. Ce groupe armé, responsable d’exactions massives, avance en territoire congolais avec des moyens militaires incompatibles avec ceux d’une simple rébellion locale. Nous avons affaire non pas à une guerre civile, mais à une agression dissimulée, aux conséquences humanitaires désastreuses. Les chiffres sont éloquents plus de 6,9 millions de déplacés internes et des milliers de civils massacrés, sans parler des violences sexuelles systématisées. Les structures de santé sont débordées, notamment à Goma, où plus de 4 500 blessés ont été pris en charge à la fin

à nommer les responsables, à agir et à peser pour mettre fin à ce conflit qui menace tout l’équilibre de l’Afrique centrale ? Envisagez vous de prendre des sanctions, comme l’ont déjà fait l’Allemagne, le Canada et d’autres nations ? La

importante de la crise se déroulant dans l’est de la RDC, qui est actuellement l’une des plus graves au monde. La diplomatie française est mobilisée sur tous les fronts pour que la paix revienne dans cette région, qui a déjà été trop meurtrie. Notre objectif est clair obtenir un cessez le feu et permettre la reprise du dialogue entre les parties. Le Président de la République et le ministre de l’Europe et des affaires étrangères sont en contact régulier avec leurs homologues de la région pour les appeler à cesser les hostilités et à reprendre le dialogue.

le droit international doit être respecté et les armes ne résoudront pas les problèmes complexes de l’est de la RDC. La France continuera de se mobiliser en ce sens. Au Conseil de sécurité de l’ONU, la diplomatie française est depuis longtemps mobilisée. Elle y a récemment défendu la résolution 2773, qui a été adoptée à l’unanimité le 21 février dernier. Celle ci condamne pour la première fois en des termes aussi clairs l’offensive du M23 et la présence rwandaise en RDC. Elle appelle le Rwanda à mettre fin à son soutien au M23 et à se retirer du territoire de la RDC. Le Conseil

Vous le voyez, nous sommes mobilisés sur tous les fronts, en soutien des médiations régionales africaines, pour que les conditions d’une paix et d’une prospérité durables dans les Kivu soient enfin réunies. La parole est à Mme Hélène Conway Mouret,

Cette situation résulte notamment du fait que les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) sont des guichets uniques recueillant toutes les demandes, qu’elles viennent de France ou du reste du monde. Si les Français vivant à l’étranger peuvent choisir n’importe quelle MDPH

par ces derniers, je vous ai proposé la création d’une MDPH qui leur serait dédiée, en concertation avec les conseillers des Français de l’étranger, dont je salue le travail et l’engagement sur ce dossier.

Monsieur le ministre, si la création d’une « MDPH 99 » ne semble pas envisagée, les besoins sont réels et les dysfonctionnements persistent, malgré les efforts des différents groupes de travail mis en place par l’AEFE et la pourquoi ne pas implanter un guichet au sein d’une MDPH existante, qui centraliserait les demandes de toutes les familles et dont les personnels seraient spécifiquement formés ? améliorerait l’accompagnement des familles et garantirait que l’école inclusive soit accessible à tous nos enfants, où qu’ils se trouvent.

afin de mieux leur faire appréhender les spécificités des demandes et des procédures propres aux Français de l’étranger en situation de handicap. Pour toute urgence ou lorsque le délai d’instruction se prolonge au delà de la moyenne, nos services – et plus spécifiquement la DFAE et les postes consulaires – saisissent la MDPH concernée en vue d’inscrire le dossier à la commission pluridisciplinaire. Pour répondre à votre question, la création d’une MDPH consacrée aux Français de l’étranger a fait l’objet d’une réflexion au sein d’un groupe de travail en lien avec la CNSA. Jusqu’à présent, cette réflexion n’a pas été conclusive, principalement en raison du nombre limité d’allocataires en situation de handicap résidant à l’étranger au regard du nombre moyen d’allocataires gérés par une MDPH en France. S’agissant des aides au financement des AESH, l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger est associée aux travaux en cours avec la CNSA en vue de faciliter les procédures pour les familles à l’étranger. Ces travaux portent notamment sur la systématisation des notifications pluriannuelles,

relative aux aspirations endotrachéales, qui entraîne des difficultés d’application pour les parents dont les enfants sont atteints de maladies rares les empêchant de s’alimenter par eux mêmes. En effet, elle prévoit que le maintien de la liberté des voies respiratoires nécessite chez les personnes trachéotomisées des aspirations endotrachéales périodiques. Ces gestes peuvent être pratiqués par les parents et, en cas d’indisponibilité, par des infirmiers ou des masseurs kinésithérapeutes habilités à les accomplir. En

Les parents sont alors obligés de s’absenter de leur travail à l’heure du déjeuner pour brancher et débrancher l’alimentation de leur enfant, y compris lorsqu’il est à l’école, car le personnel scolaire n’est pas autorisé à faire ce geste. À ce jour, de nombreux parents sont concernés par le manque de disponibilité de tiers susceptibles d’assurer périodiquement périodiquement et très rapidement ces aspirations endotrachéales. Il a même été constaté que, dans certains instituts médico éducatifs (IME), les infirmières responsables des enfants trachéotomisés

très rapidement. Les patients qui ont l’usage de leurs mains les réalisent eux mêmes. Lorsque ce n’est pas le cas, ils doivent avoir recours à l’assistance d’un tiers. Jusqu’en 1999, seuls les infirmiers et les masseurs kinésithérapeutes étaient habilités à à accomplir ce geste, ce qui compromettait le retour à domicile ou l’accueil en structure d’hébergement de personnes dont l’état ne nécessitait plus une hospitalisation et posait problème aux parents ayant des enfants à la maison.

dont la mise en œuvre est prévue pour le 1 janvier 2026, suscite de nombreuses inquiétudes chez les professionnels de la petite enfance.

ce qui menace directement l’avenir du secteur de la petite enfance. En effet, les nouvelles normes pourraient entraîner la disparition de 80 000 places d’accueil et la fermeture de plusieurs milliers de microcrèches sur l’ensemble du territoire français, alors même qu’il existe déjà une pénurie de professionnels qualifiés dans ce secteur. Madame la ministre, ma question s’articule en deux temps. Pouvez vous nous confirmer que cette réforme ne s’appliquera pas aux 15 000 professionnels déjà en poste qui sont titulaires d’un CAP petite enfance et que le niveau de qualification exigé ne s’appliquera aux recrutements qu’à compter du 1 septembre 2026 ? Par ailleurs, vous engagez vous à entamer un processus de concertation sur le calendrier de déploiement de cette réforme, sur la formation de professionnels en urgence pour répondre aux nouvelles exigences de qualification et sur la mise en œuvre de mesures transitoires ?

ce projet de décret, qui vient d’être examiné par le Conseil d’État. Il a pour objet d’aligner les normes d’encadrement des microcrèches sur celles des crèches classiques de taille similaire, les petites crèches. Ainsi, les microcrèches devront compter au moins

Les auxiliaires de puériculture ou tout autre professionnel occupant le poste de référent technique avant cette date pourront être maintenus à leur poste. poste. Les titulaires d’un CAP présents dans les crèches n’auront pas à acquérir le diplôme d’État d’auxiliaire de puériculture et pourront continuer d’exercer. En effet, de

essentielles pour respecter les besoins des enfants et assurer leur sécurité. En effet, les enfants accueillis dans les microcrèches étant les mêmes que ceux qui sont accueillis dans les petites crèches classiques, il n’y a aucune raison que les conditions d’encadrement diffèrent.

de l’autonomie et du handicap. Madame la ministre, en France, plus de 11 millions de personnes soutiennent un proche en situation de handicap, de perte d’autonomie ou de maladie chronique ou invalidante.

Elle déplorait, d’une part, le peu d’appels à projet ou à manifestation d’intérêt et, d’autre part, la réticence des ARS à financer ce type d’offre, qui tient de l’expérimentation. Pourtant, la création de résidences de répit partagé aidés aidants offre une solution innovante, dont les nombreux atouts ont déjà été longuement évoqués dans cet hémicycle.

et notamment des solutions de répit pour les familles. Sur le terrain, cette hausse des moyens est attendue par les ARS et par les porteurs de projet. Je pense en particulier au projet expérimental ciblé sur la commune de Luxeuil les Bains, dans le département de la Haute Saône, qui présente la particularité médicale de permettre l’accès des aidants aux soins thermaux. Madame la ministre, confirmez vous que cette enveloppe de 80 millions d’euros servira

les domaines de leur vie : leur santé, leur activité professionnelle, leur bien être, leur temps libre. Aussi, ils expriment un besoin de répit, notamment lorsque le proche qu’ils aident vit à leur domicile.

Chacun le sait, les entreprises ont recours aux contrats d’apprentissage pour recruter à un coût significativement moins élevé que celui de le cap du million de jeunes en apprentissage a été franchi l’an dernier, l’augmentation du reste à charge risque d’entraîner une baisse substantielle du nombre d’apprentis, en raison d’une perte d’attractivité économique. Un tel retour en arrière serait

les représentants des branches professionnelles et les partenaires sociaux. Il s’agit de redonner la main aux branches professionnelles pour qu’elles puissent décider d’elles mêmes de variations beaucoup plus fortes sur les coûts contrats

Si l’on ajoute à cela l’absence de consultation des conseils départementaux et la non prise en compte des propositions de Départements de France, nous réunissons tous les ingrédients d’une réforme mal engagée, dont le calendrier précipité et le manque de discussions préalables risquent de rendre difficile le déploiement.

Enfin, à la demande de Départements de France, un comité mensuel de suivi de la réforme a été installé. Il s’est réuni pour la première fois vendredi dernier.

Cet axe autoroutier est un corridor stratégique, tant pour le trafic que pour la sécurité des usagers. Il semble difficilement compréhensible que cette inertie bloque une décision de bon sens, attendue par tous les acteurs de terrain pour une meilleure efficacité de l’action publique. Madame la ministre, le Gouvernement entend il clarifier la situation en actant rapidement ce transfert, afin de garantir une gestion cohérente et efficace de la sécurité sur cette portion de l’A1 ? La parole est

Comme vous le précisez, la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 dispose que les sapeurs pompiers volontaires ayant accompli plus de dix ans de service peuvent bénéficier de trimestres de retraite selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

en janvier dernier. Chaque année, près de 6 000 communes font l’objet d’une reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, en grande majorité à cause d’inondations. À elles seules, ces dernières entraînent des indemnisations annuelles de l’ordre de 20 milliards d’euros, selon les services du Gouvernement, qui ne prennent pas en compte les indemnisations versées pour les véhicules sinistrés. À titre d’exemple, les dommages subis cette année par le magasin Leclerc de Saint Nicolas de Redon sont estimés à 9 millions d’euros, auxquels s’ajoutent 6 millions d’euros pour les commerces de la galerie marchande. ces coûts sont lourds de conséquences. En 2021, notre collègue Jean Yves Roux alertait déjà vos prédécesseurs quant aux réticences des compagnies d’assurances à couvrir les équipements publics des communes, du fait des risques climatiques. Ce frein risque fort d’être étendu aux entreprises et aux particuliers victimes d’inondations. Or, pour bénéficier des dispositifs mis en œuvre en cas de reconnaissance de catastrophe naturelle, il faut être couvert par un contrat d’assurance. Dès lors, quelles pistes envisagez vous pour garantir aux communes, aux entreprises et aux habitants des indemnisations à la hauteur des dégâts subis lors des inondations ?

ou des contrats automobiles. Au total, le régime d’indemnisation des catastrophes naturelles disposera ainsi d’une capacité de couverture supplémentaire de 1,2 milliard d’euros par an.

Dans des territoires où l’offre de transports en commun est souvent inexistante, ne pouvoir conduire signifie être isolé, éloigné des opportunités professionnelles et limité dans son quotidien.

mer et de la pêche. Madame la ministre, les filières à responsabilité élargie du producteur (REP) partent du principe selon lequel les producteurs sont responsables du financement ou de l’organisation de la prévention et de la gestion des déchets issue des produits en fin de vie.

Depuis plusieurs mois déjà, les professionnels, auxquels je me suis joint, alertent quant au risque réel de déstabilisation de l’ensemble de cette filière. En effet, les filières REP font face à des prises de marges successives et cumulatives sur le montant de l’écocontribution. Ces prises de marges augmentent artificiellement les prix des produits. Elles conduisent aujourd’hui certains professionnels à remettre en cause le versement des écocontributions. Aussi est il urgent de pérenniser le principe de non réfaction et de répercussion à l’identique de l’écocontribution de la REP ameublement et de généraliser ce principe à l’ensemble des filières ; je pense notamment à la filière des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment. Madame la ministre, allez vous répondre à cette demande ?

ainsi incités à améliorer l’écoconception. Les producteurs concernés s’acquittent généralement de leurs obligations en mettant en place collectivement des éco organismes auxquels ils transfèrent leurs obligations. Ils versent, en contrepartie, une contribution financière. Dans la filière des équipements électriques électroniques comme dans la filière des meubles, cette contribution visible a été mise en place selon des modalités particulières, visant à la répercuter jusqu’au consommateur final.

tout en réduisant l’intensité concurrentielle. De telles dispositions présentent à la fois des avantages et des inconvénients. Il convient de les évaluer au regard de l’intérêt que peut présenter le dispositif

particulière à ce phénomène, parce qu’il a des conséquences économiques graves. Une indemnisation des pertes, directes

30 % en février 2024. Il est aussi prévu une indemnisation pour les femelles gestantes ou reproductrices à une valeur de près de deux à cinq fois plus élevée que celle des agneaux, pour tenir compte de ce potentiel reproducteur.

Ce dossier, baptisé Parc éolien de la Tonnelle, se situe sur le territoire de la communauté de communes Gâtinais Val de Loing et concerne les communes de Souppes sur Loing, de Poligny et de Bagneaux sur Loing.

Dans le cadre de sa compétence en matière d’environnement, la communauté de communes s’inscrit déjà fortement dans plusieurs projets liés aux énergies renouvelables et prend sa part dans l’introduction d’énergies propres. Ainsi, parmi d’autres installations, 25 éoliennes sont d’ores et déjà en place. La communauté de communes Gâtinais Val de Loing et les communes incluses dans la zone d’implantation potentielle (ZIP) ont fait part de leur opposition au projet, alors que la concertation est ouverte depuis le 5 février 2025. Le tracé a été réalisé en respectant plusieurs contraintes posées par les services de l’État et les gestionnaires de réseaux, mais la voix des collectivités doit être entendue. La procédure de concertation a été placée sous l’égide de la Commission nationale du débat public Une demande d’autorisation environnementale devra être déposée à son issue. Ma question est simple, madame la ministre : quelle est la position du Gouvernement sur ce projet ?

S’il vise principalement des pays comme l’Indonésie, il omet totalement la réalité guyanaise. Ainsi, la Guyane couverte à plus de 96 % par la forêt, dont 95 % de forêt primaire, en sera une victime collatérale.

En effet, la Guyane est la seule région française dont la surface agricole utile connaît une croissance continue, pour répondre à la forte augmentation démographique et au défi de la souveraineté alimentaire, prônée par l’État.

le Gouvernement doit agir vite et fort et demander pour la Guyane une dérogation à l’application de ce règlement. Il y va du développement de la Guyane, de son agriculture et de sa capacité à bâtir un avenir durable pour ses habitants. Après l’interdiction des forages pétroliers, les difficultés que rencontrent les orpailleurs légaux, le blocage des aides aux pêcheurs, maintenant, nous en arrivons à

à laisser entrer sur le marché de l’Union européenne et à permettre l’exportation de certains produits de base ou associés à la déforestation et à la dégradation

à certains espaces une vocation agricole, visant, comme vous l’avez évoqué, le développement économique et l’autonomie alimentaire de la région.

au mois d’octobre dernier, le directeur de la prison de Majicavo démissionnait pour dénoncer la situation de surpopulation carcérale, laquelle de plus en plus de tensions entre les détenus et le personnel pénitentiaire. Ce dernier a été éprouvé par la mutinerie du 28 septembre 2024. Le taux d’occupation élevé, puisqu’on y compte 650 détenus pour 278 places. Cette surpopulation carcérale est aggravée par un manque d’infrastructures judiciaires et carcérales essentielles pour la vie d’un département

Le 28 octobre 2024, il m’a répondu que la planification de la construction des infrastructures judiciaires me serait rapidement communiquée. Je n’ai à ce jour pas d’autre réponse. Je vous demande donc, madame la ministre, de m’indiquer la programmation des investissements, avec calendrier, des infrastructures judiciaires que je viens de mentionner.

dont la situation est encore difficile, ainsi qu’aux personnels du ministère de la justice qui, sur place, assurent avec courage et résilience

Un premier terrain a été identifié pour l’accueillir, à proximité du centre de Mamoudzou. Le démarrage de la phase d’études est prévu en 2026. Afin d’améliorer les conditions de travail des personnels pénitentiaires et la prise en charge des personnes détenues, la construction d’un second centre pénitentiaire à Mayotte a été annoncée en 2022, sur la base d’un projet de construction de 400 nouvelles places de détention. En mars 2023, En mars 2023, comme vous le savez, des recherches foncières ont commencé. Le garde des sceaux a demandé à ses services de se rendre sur place très prochainement,

et de la recherche. Madame la ministre, ma question concerne les écoles parisiennes. En effet, communauté scolaire parisienne est en colère depuis de nombreuses semaines, de nombreux mois.

compte t il revenir sur ces suppressions de postes, notamment dans les zones situées en REP ?

est, de manière générale, sensible sur tous les territoires, particulièrement à cette époque de l’année. Il l’est aussi, naturellement, dans l’académie de Paris, où la baisse démographique, qui nous touche tous, sera particulièrement sensible à la rentrée prochaine,

ce nombre est de 20, donc inférieur. La lutte contre les inégalités sociales, que vous évoquez, est aussi notre priorité. Mais à Paris, en éducation prioritaire, 8 élèves sur 10, tous niveaux confondus, sont scolarisés dans des classes de moins de 20 élèves. Les fermetures prévues se traduiront donc, non pas par une baisse, mais par une hausse du taux d’encadrement. Nous y sommes attentifs. Par ailleurs, les directeurs des écoles publiques de Paris bénéficient d’un régime dérogatoire de décharges d’enseignement. Depuis 1982, les directeurs des écoles parisiennes sont ainsi déchargés de leurs fonctions d’enseignement, se consacrant totalement

En septembre, la Cour des comptes a pointé du doigt cet état de fait et a demandé au Gouvernement d’y mettre fin. Le ministère a donc lancé une concertation avec la Ville.

Les passagers devront donc encore subir, pendant trois ans, des locomotives de plus de 40 ans et des voitures Corail à bout de souffle, qui connaissent de nombreuses pannes, malgré le travail sérieux des cheminots. S’agissant du trafic,

cette ligne ferroviaire, stratégique, dessert 4 régions, 32 départements et 5 millions d’usagers potentiels. Au cœur de la ligne se situe, Gaillarde, une étoile ferroviaire stratégique pour les départements de la Corrèze, du Lot, de la Dordogne, du Cantal et de l’Aveyron. Elle doit être protégée. Madame la ministre, il est essentiel d’écouter et de prendre en compte la voix des territoires ruraux, des villes moyennes et des entreprises. Quelles solutions concrètes

depuis 2023, de plus en plus de collectivités territoriales ont subi la résiliation unilatérale de leur contrat de la part de leur assureur. Plusieurs propositions ont été formulées pour lutter contre le phénomène

Ma question est simple : envisagez vous des ajustements ou des dérogations pour que ces communes bénéficient enfin du soutien auquel elles peuvent légitimement prétendre ?

Cette annonce ne fut précédée d’aucune information ou consultation préalable avec les acteurs publics et privés du département de la Creuse. Elle révèle un manque patent d’anticipation du gestionnaire et survient après d’autres décisions analogues : je pense à la fermeture de la ligne Ussel Montluçon, qui desservait jusqu’en 2008 toute la partie est du département. La mort programmée de cette ligne de désenclavement reliant la préfecture de Guéret à la sous préfecture d’Aubusson est désastreuse en matière de service à la population, de développement économique,

français, et empêche de rejoindre Bordeaux, capitale régionale, Limoges. Les besoins de régénération de la voie sont urgents et indispensables à la sécurisation de la circulation et à la pérennisation de la ligne. Il est de la responsabilité de l’État, de la région Nouvelle Aquitaine et de la SNCF de trouver les moyens de financer sa sauvegarde. Le succès remporté par la pétition « Touche pas à ma p’tite ligne ! », qui a recueilli près de 25 000 signatures, traduit le profond attachement des élus et de la population locale à cette desserte fine du territoire. confirme la nécessité de préserver le ferroviaire, qui demeure la mobilité la plus décarbonée et la mieux adaptée à la lutte contre le réchauffement climatique. Que comptez vous faire concrètement pour assurer le maintien en service et la rénovation de cette liaison autour de dessertes suffisamment cadencées et d’une tarification attractive ? Quelle garantie êtes vous en mesure d’apporter pour mettre un terme à cette fracture ferroviaire qui éprouve ce département ? La

le maintien, la préservation et la remise en état des petites lignes ferroviaires. En 2021, un protocole a été signé entre l’État et la région Nouvelle Aquitaine pour déterminer

est à la charge du conseil régional de Nouvelle Aquitaine. Les études conduites dans le cadre du contrat de plan État région (CPER) 2023 2027 ont permis d’identifier un besoin de travaux d’urgence, d’un montant

toutes les solutions de mobilité envisageables afin de maintenir cette liaison essentielle pour les habitants de la Creuse, en concertation avec l’ensemble des acteurs concernés. La réflexion sur l’avenir de cette ligne a été inscrite au deuxième plan particulier pour la Creuse (PPC2), qui devrait être bientôt

les aménagements votés dans le cadre de la loi de finances pour 2025. Sur les 43 communes qui composent l’intercommunalité, 21 communes du bassin de vie de Marmande sont actuellement exclues du dispositif.

des médecins partent et des entreprises délocalisent leurs activités à quelques kilomètres pour bénéficier de la fiscalité propre aux zones FRR. Ces mouvements de dumping fiscal réorganisent l’espace et les activités dans un territoire déjà fragilisé par le chômage et un taux de pauvreté important.

Si le déclassement devait perdurer, Marmande pâtirait à coup sûr de cette situation d’isolement fiscal, ce qui nuirait à son attractivité et à son dynamisme. Je suis certain que ce n’est pas l’objectif visé par le Gouvernement. Madame la ministre, pouvons nous envisager ensemble le réexamen rapide de ce dossier ? La parole est

recueilli leur avis. Ce tronçon fait partie du Grand Genève et constitue, avec 50 000 véhicules par jour, une autoroute urbaine de contournement.

Au delà du strict impact financier, notamment pour les milliers de salariés payés en euros qui utilisent quotidiennement ce tronçon et qui sont les premières victimes de l’augmentation du coût de la vie dans le département, cette décision unilatérale de l’État risque d’entraîner un report massif du trafic sur le réseau secondaire, déjà fortement saturé. Ce renvoi de circulation route départementale (RD) 1206, va inévitablement créer des nuisances environnementales et sonores pour des milliers de riverains déjà bien éprouvés par le ballet incessant de véhicules en provenance ou à destination de la Suisse voisine.

saluer votre engagement. Vous posez la question des conséquences de la régularisation des péages qui concernent la section de l’A40 entre Annemasse et Saint Julien en Genevois.

du doigt par la Cour des comptes en 2019. Le Gouvernement a souhaité prendre le temps de la concertation pour régulariser la question du péage sur cette section

paieront moins de 1 euro le trajet entre Annemasse et Saint Julien en Genevois. Par ailleurs, les conditions de circulation des usagers seront améliorées par des aménagements réalisés aux deux extrémités de la section, au niveau de Saint Julien en Genevois et d’Étrembières.

sera consacrée à l’accompagnement des aménagements qui pourraient être entrepris par les gestionnaires sur le réseau secondaire, en lien avec l’opération. La parole madame la ministre : vous savez autant que moi que ces mesures compensatoires ne suffiront pas à nous faire avaler la pilule ! Aucune raison financière ne justifie la fin de cette gratuité, car la société concessionnaire est largement bénéficiaire. Bien sûr ! Nous faisons

percutés par un train alors que leur véhicule traversait un passage à niveau. Permettez moi d’avoir une pensée pour leurs familles, leurs frères d’armes et les blessés. Ce drame vient s’ajouter à la longue liste des accidents survenus à des intersections critiques entre la route et le rail. Malgré les efforts de sécurisation engagés depuis plusieurs années, les passages à niveau restent un véritable danger sur notre réseau routier. d’entre eux ont été supprimés ou modernisés, mais force est de constater que trop peu de moyens sont alloués pour améliorer significativement la situation. Les collectivités locales, qui sont en première ligne pour assurer la sécurité des infrastructures, peinent à obtenir les financements nécessaires. Les infrastructures vieillissantes nécessitent pourtant une modernisation urgente et leur sécurisation doit être une priorité absolue. Les communes et départements, qui disposent souvent de budgets contraints, ne peuvent pas assumer seuls les investissements colossaux nécessaires à la mise en conformité de ces équipements.

Face à cette réalité, il est urgent que l’État prenne ses responsabilités et accompagne bien plus activement les collectivités locales dans la modernisation et la sécurisation des passages à niveau. Cela passe bien évidemment par une augmentation significative des crédits afférents, mais aussi par une simplification des démarches administratives, qui freinent trop souvent la mise en œuvre des projets. Madame la ministre, quelles mesures concrètes votre gouvernement compte t il prendre pour renforcer cet accompagnement ? Quels nouveaux financements seront mobilisés pour aider les collectivités à supprimer ou moderniser les passages à niveau les plus dangereux ? Enfin, pouvez vous nous garantir que la sécurisation de ces infrastructures deviendra une véritable priorité, pour éviter que de telles tragédies ne se reproduisent encore et protéger nos concitoyens d’un danger qui ne devrait pas en être un ? La parole

millions d’euros dans le cadre du plan de relance. Je tiens à vous assurer que les crédits de l’État disponibles en 2025 pour la sécurisation des passages à niveau permettent de couvrir les besoins exprimés par les préfets de région. Je vous confirme que le Gouvernement est déterminé à poursuivre ses efforts pour que des drames comme celui de Bailleul Sir Berthoult ne se reproduisent plus.

Chacun peut constater que la durée des procédures et des recours devient un frein non négligeable. De plus, la motivation des décisions n’est souvent pas de nature à rendre compréhensibles les choix opérés. Notons également le sentiment d’injustice frappant les jeunes agriculteurs, qui voient des fonciers rétrocédés à des agriculteurs déjà installés. sentiment est d’autant plus prononcé lorsqu’il est fait recours à des prête noms ou des sociétés opaques. La durée des recours devient intolérable. Cette situation semble être en partie due au mode de fonctionnement des Safer et des moyens financiers dont ces établissements publics disposent. Mis en place en 1960, ces outils sont nécessaires, mais ils doivent impérativement s’adapter, étant donné les évolutions importantes que connaît le secteur de l’agriculture et le rôle fondamental joué par les agriculteurs dans l’économie française.

est à Mme la ministre. Madame la sénatrice Marie Claude Lermytte, je partage votre préoccupation pour l’installation des jeunes agriculteurs. Le renouvellement des générations en agriculture est un défi majeur

propice à la réalisation d’opérations complexes. En outre, cela laisse du temps aux acquéreurs pour parfaire leur dossier et permet aux jeunes agriculteurs d’obtenir des garanties bancaires pour leur projet. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement appuie fortement toutes les options de transmission du foncier agricole hors acquisition.

l’acquisition est ainsi retardée, au moment où l’exploitation est financièrement stabilisée. Par ailleurs, les commissaires du Gouvernement auprès des Safer, qui relèvent à la fois du ministère de l’agriculture et du ministère des finances, exercent une tutelle appuyée sur ces en vue notamment d’obtenir des éléments clairs, précis et non stéréotypés sur la motivation des décisions de rétrocession. C’est un point central pour assurer l’intelligibilité et l’acceptabilité des décisions.

Or cette absence de reconnaissance officielle est en contradiction complète avec les observations récurrentes et documentées sur le terrain. C’est pourquoi, madame la ministre, au regard de ces éléments, je vous demande de préciser les critères et la méthodologie utilisés par l’OFB pour cartographier la présence du loup.

La méthode d’estimation de la population du loup a fait l’objet d’une évolution en 2024, pour trois raisons. Premièrement, l’OFB publiait jusqu’alors deux chiffres par an et il a été décidé de disposer d’une estimation unique pour une meilleure lisibilité deuxièmement, les marges d’erreur de l’ancienne méthodologie étaient de plus en plus importantes, ce qui ruinait la confiance à l’égard des chiffres et nourrissait la colère des éleveurs troisièmement, vous admettrez qu’il existait un réel besoin de transparence. La nouvelle méthode, basée sur les données génétiques, a été présentée aux membres du groupe national Loup à la fin de l’année 2024, pour une mise en œuvre en 2025. Je peux vous assurer que, grâce au travail de l’OFB,

les efforts de l’OFB portent sur une meilleure répartition de la collecte des indices afin d’assurer un suivi homogène. Pour cela, l’Office a développé une carte accessible au grand public sur le site. Vous Vous pourrez y retrouver les indices recueillis pour la Nièvre et le traitement qui leur a été réservé. Cela apporte un gage de transparence essentiel dans ce dossier.

Au fil des années, cela permettra de mieux comprendre comment les loups se répartissent, de mieux réguler leur présence et ainsi de mieux répondre aux attaques qu’ils opèrent sur nos élevages. Il faut conclure. Tel est le vœu que je forme et je peux vous assurer, madame la sénatrice, que j’y porterai une attention toute particulière.

de la souveraineté alimentaire. Madame la ministre, les producteurs d’œufs traversent une crise majeure. Actuellement, dès qu’un prélèvement unique détecte une suspicion de salmonelle, tout le cheptel doit être abattu. abattu. Or ces résultats sont souvent discutables et des analyses complémentaires réalisées par des laboratoires accrédités montrent régulièrement qu’il n’existe en réalité aucune contamination. Ce système est un véritable désastre pour les éleveurs. En un an, le cheptel de poules pondeuses en Alsace a chuté de 17 %, soit plus de 175 000 volailles en moins. Certains exploitants sont à bout.

rapidement : ajouter un second test de confirmation avant l’abattage, comme cela se pratique déjà en Belgique et aux Pays Bas, Bas, tester directement les œufs destinés à la consommation, car c’est là que se situe le véritable risque pour le consommateur, plutôt que d’analyser des poussières ou des fientes, ou encore assouplir les règles quand les œufs sont destinés à être consommés après un traitement thermique. travail (Anses), saisie depuis le début de 2023 pour revoir ses procédures, n’a toujours pas rendu ses conclusions. Il est donc urgent de savoir quelles mesures seront prises pour répondre aux attentes des éleveurs et éviter l’effondrement de cette filière essentielle.

dont l’enjeu est important pour la santé publique, mais aussi pour la filière des ovoproduits. Les méthodes de prélèvement en élevage sont basées sur les caractéristiques propres des salmonelles.

Concernant les résultats d’analyse, j’attire votre attention sur le fait qu’ils émanent de laboratoires agréés soumis à des essais interlaboratoires, supervisés par le laboratoire national de référence. Ils sont donc particulièrement fiables. Par ailleurs, mon ministère a saisi l’Anses sur l’optimisation des méthodes actuelles de prélèvement en élevage. Une étude est en cours et la restitution des travaux aura lieu au début de l’automne 2025. Pour ce qui est de l’impact économique,

Enfin, d’un point de vue de santé publique, les salmonelles présentes sur les viandes de volaille peuvent être tout aussi dangereuses que celles qui se trouvent dans les œufs. Ainsi, la viande de volaille issue d’animaux contaminés par une salmonelle peut s’avérer extrêmement dangereuse, soit en raison d’une cuisson incomplète, parfois sous l’effet de nouveaux modes de consommation, soit à la suite d’une contamination croisée lors de la préparation des repas. des repas. De telles situations sont susceptibles de provoquer des salmonelloses chez le consommateur. Il nous faut donc tout mettre en œuvre pour préserver la santé humaine, mais aussi la confiance dans les produits et ainsi assurer la pérennité de nos filières. La parole

et de la souveraineté alimentaire. Déjà fragilisé par la concurrence étrangère et par des prix de vente des animaux insuffisants, l’élevage français fait désormais face à une accumulation de périls sanitaires.

suite des alertes des éleveurs et des parlementaires, votre ministère a réagi en urgence : 14 millions de doses de vaccins contre la FCO ont été commandées l’an dernier et des avances d’indemnisation ont été versées sur la base des déclarations des éleveurs. Ces efforts de vaccination et de simplification administrative doivent évidemment être salués ils ont permis de réduire la mortalité et de sauver la trésorerie de milliers d’exploitations. Pour autant, cette réponse est incomplète, car les vaccins manquent toujours et la France est encore dépendante d’importations pour se les procurer. Surtout, il nous faut nous préparer aux futures épidémies, qui vont se multiplier dans les années à venir. Le réchauffement climatique et les échanges internationaux entraînent l’arrivée de nouvelles maladies auxquelles nous sommes très peu préparés, comme la FCO et ses différents variants ou la Ces nouvelles maladies requièrent une véritable anticipation, une planification, une coordination, une adaptation, et les éleveurs attendent à ce titre des réponses de l’État. Vous avez lancé les assises du sanitaire animal. Quel en est le périmètre ? Au vu de l’urgence, quelles mesures allez vous prendre dès maintenant pour garantir la disponibilité des vaccins ? Par ailleurs, alors que de nouvelles souches de virus pour lesquelles nous n’avons pas de vaccins apparaissent, comme la FCO 12 aux Pays Bas, quels moyens allez vous mettre en œuvre pour renforcer la recherche scientifique, les services vétérinaires et l’équarrissage ? Enfin, comment allez vous prendre en compte les spécificités de l’élevage en plein air,

vous me posez une question légitime à laquelle je n’ai eu de cesse de répondre avec le Gouvernement depuis le premier jour de mon arrivée au ministère, depuis le premier jour de la crise sanitaire qui touche le cheptel français. Je vous remercie à ce titre d’avoir rappelé les différentes mesures que nous avons mises en place. Du 2 août 2024 au 16 février 2025, une zone régulée a été créée afin de limiter l’extension de la maladie et de préserver les échanges commerciaux avec les autres États membres. Dès le printemps 2024, une ambitieuse campagne de vaccination a été déployée sur l’ensemble du territoire, effective à partir du mois d’août 2024. L’État a passé commande de 14 millions de doses de vaccins, pour un montant de 37 millions d’euros, afin de réduire les conséquences sanitaires sur les cheptels. En dépit d’un contexte budgétaire défavorable, j’ai mis en place dès mon arrivée au Gouvernement, avec l’accord du Premier ministre de l’époque, un fonds d’urgence exceptionnel de 75 millions d’euros, qui a permis de répondre à l’intégralité des demandes d’indemnisation déposées. Par ailleurs, le Gouvernement a tenu son engagement de réactivité pour aider les éleveurs en déployant deux guichets : un guichet « avance », qui a permis de répondre à l’urgence en novembre 2024 à hauteur de 30

Au delà de ces réponses en urgence, je suis convaincue qu’une stratégie sanitaire résiliente, axée sur l’anticipation et la prévention des maladies, est nécessaire. C’est pourquoi j’ai lancé les assises du sanitaire animal le 30 janvier dernier, dont j’ai présidé la réunion de lancement devant plus de 200 acteurs du sanitaire et des professionnels de l’élevage. L’année 2025 sera donc une année de transition, pour laisser le temps aux filières et au ministère de l’agriculture de coconstruire les contrats sanitaires de filières. J’ai demandé à chacune d’entre elles d’élaborer le sien et nous travaillons

et face à l’insuffisance des capacités d’équarrissage, l’État a ouvert en urgence plusieurs sites d’enfouissement. Une zone de préstockage temporaire sous contrôle devant accueillir les cadavres de volailles est alors créée sur la commune de Petosse, en Vendée. Cette installation s’est faite sans que les élus locaux en soient informés en amont. Huit mois plus tard, en décembre 2022, la fosse a récupéré les restes du site de Tallud Sainte Gemme, fermé en raison de risques de ruissellement.

Madame la ministre, vous n’étiez alors pas en responsabilité, mais il est important de rappeler que le maire et les habitants ont subi cette situation sans explications ni anticipation et que cette fosse aurait dû fermer il y a déjà un an : sa durée d’exploitation était fixée à vingt quatre mois. Pourtant, près de 13 700 tonnes de matières solides y sont encore stockées, en dépit des engagements pris. Pendant des mois, les élus locaux ont été laissés sans soutien ni réponse à leurs sollicitations. Jusqu’à récemment, aucune information ne leur avait été communiquée sur les résultats des tests sanitaires réalisés. Un rapport d’inspection préparé en début d’année énumère plusieurs solutions pour vider cette fosse. Malgré ces propositions, les modalités de traitement et d’évacuation des matières stockées n’ont pas été tranchées. Madame la ministre, quelle solution le Gouvernement entend il retenir pour résoudre cette situation ? Surtout, dans quel délai compte t il la mettre en œuvre ? La parole est à Mme la ministre. est à Mme la ministre. Madame la sénatrice Annick Billon, vous posez une question légitime et le Gouvernement est conscient des enjeux autour de ce site de stockage temporaire de cadavres de volailles de Petosse. Permettez moi de rappeler que la France a fait face entre 2019 et 2023 à plusieurs épidémies d’influenza aviaire dans les élevages de volailles. En mars 2022,

deux sites temporaires de stockage de cadavres sur les communes de Tallud Sainte Gemme et de Petosse, dans votre département. Afin d’assurer la maîtrise des risques sanitaires et environnementaux, ces mesures ont été prises de manière concertée entre les différents services des ministères chargés

dans le cadre d’une gestion de crise. Sa qualité a d’ailleurs été saluée par les représentants de la Commission européenne, venus constater la gestion globale de la crise de l’influenza aviaire

afin de définir les options possibles quant au devenir des matières stockées, les dispositifs d’évacuation et le processus de restitution du terrain. Son rapport vient de m’être présenté. Mon cabinet et les services en examinent les conclusions et les recommandations. Je prendrai donc une décision dans les mois à venir, conformément aux recommandations de ce rapport et en collaboration avec les autorités locales, dont vous êtes. La parole

de la tarification de l’eau entrée en vigueur le 1 janvier 2025 pour les agriculteurs irrigants raccordés au réseau d’eau potable. Assujettis, comme l’ensemble des usagers, à une redevance pour consommation atteignant 0,43 euro par mètre cube dans les Alpes Maritimes, ces professionnels maralpins, dont près de 80 % sont raccordés pour subvenir aux besoins d’une agriculture à taille humaine, sobre en intrants et orientée vers le maraîchage multirotation, font état d’une situation financièrement intenable. Les factures reçues en 2025 et portant sur les consommations de 2024 intègrent déjà la nouvelle redevance. Cette charge, mise en œuvre sans concertation préalable et pesant de manière disproportionnée sur les secteurs agricole et agroalimentaire, est particulièrement inquiétante dans mon département, où les agriculteurs sont placés dans un état contraint de dépendance au réseau d’eau potable. Cette situation est le fruit malheureux du démantèlement des réseaux agricoles, de la forte pression urbaine et de l’absence d’un tarif spécifique agricole, qui aurait pour effet d’éviter la multiplication par dix des redevances actuellement appliquées aux usagers. Sans une action urgente, nous pouvons craindre des cessations d’activité en cascade ainsi que des renoncements à l’installation de de nouveaux agriculteurs. Madame la ministre, les agriculteurs maralpins ne peuvent faire face à ces hausses qui les étranglent et encore moins attendre le prochain budget. Ils aspirent à une solution rapide : la mise en suspens immédiate des factures des prestations destinées aux abonnés bénéficiant d’un compteur au sein des exploitations fortement touchées et la mise en place de dispositifs d’aide ciblés répondant aux professionnels en situation de dépendance. Pouvez vous nous éclairer sur vos intentions et sur celles du Gouvernement en la matière ?

d’un enjeu majeur pour les agriculteurs irrigants raccordés à l’eau potable, particulièrement dans votre département des Alpes Maritimes. Pour rappel, la réforme adoptée en loi de finances pour 2024 a pour objectif de rééquilibrer la contribution des différentes catégories d’usagers au financement de la politique de l’eau, de promouvoir un usage plus sobre et plus performant de cette ressource et d’améliorer la lisibilité de la fiscalité y afférente. Cet objectif de lisibilité et de simplicité se traduit par la modification des assiettes de la redevance. Les redevances de consommation d’eau potable et de performance du service d’eau potable sont assises sur la consommation ; la la redevance de performance assainissement est, quant à elle, assise sur l’eau usée rejetée au réseau d’assainissement collectif. Cela explique des hausses significatives, avec une multiplication supérieure à par rapport au régime antérieur pour un nombre important de professionnels, ce qui les met en situation de fragilité. C’est vrai pour les agriculteurs, mais aussi pour le secteur agroalimentaire, qui est très affecté.

Nous travaillons sur ce sujet avec mes collègues chargés de l’écologie, de l’industrie et du budget. Enfin, je souhaite mentionner qu’il a été donné instruction aux agences de l’eau de mettre à profit la période pour accompagner de manière proactive les industriels concernés dans la mise en œuvre de procédés plus sobres en eau potable. Tout le

d’usines en 2024, mais vous intégrez dans votre calcul les extensions de sites déjà existants, quel que soit le montant de l’investissement concerné. Or nos industries sont loin de tourner à leur pleine capacité. En décembre dernier, le taux d’utilisation des usines est tombé à 73,9

pour en bénéficier, il nous faudra survivre jusque là ! » Très franchement, si vous ne corrigez pas le tir, nous allons droit dans le mur. Je vous ai interpellée à de nombreuses reprises. Pour le moment, je n’ai pas obtenu de réponse concrète à mes questions. Quelle est la stratégie de l’État en matière de planification ?

pays. Les territoires concernés par ce tracé abritent de plus des sites naturels protégés, des monuments patrimoniaux et des paysages où se développent des activités touristiques. La construction de cette ligne pourrait ainsi menacer des emplois et fragiliser certaines entreprises locales.

Cette alternative consiste à déplacer la production d’hydrogène à Aramon, à proximité des sources d’électricité existantes, et à l’acheminer par des ouvrages enterrés le long des digues du Rhône. Cette solution garantirait une meilleure acceptabilité du projet tout en évitant la construction d’une ligne aérienne à très haute tension.

de l’industrie et de l’énergie. Dans un communiqué de presse en date du 12 février dernier, le Gouvernement a annoncé mettre en consultation un projet d’arrêté modifiant le soutien au développement du photovoltaïque sur bâtiment, hangar et ombrière.

J’ai ainsi été alerté par une entreprise de mon département qui emploie environ trente cinq salariés et qui s’alarme des conséquences des revirements incessants des décisions publiques. En avril 2024, les acteurs du secteur avaient en effet signé avec l’État un Pacte solaire, promesse d’un soutien ferme. C’était il y a moins d’un an.

facilitent la rénovation et la modernisation du patrimoine public ainsi que le financement d’infrastructures. Ne craignez vous pas que ces évolutions annoncées soient synonymes de moratoire pour les filières, madame la ministre ? En avez vous évalué les conséquences ? Par ailleurs, dans quelle mesure allez vous tenir compte des demandes de modifications formulées par le Conseil supérieur de l’énergie

la viabilité de nombreuses entreprises et la pérennité des emplois y afférents. Le photovoltaïque est une technologie mature, compétitive ; il constitue l’une des solutions les plus agiles pour réussir la transition écologique. C’est aussi une filière dynamique qui emporte l’implantation dans

2050, il n’est plus possible de faire du. Il y a moins d’un an, l’État signait avec la filière le Pacte solaire ; or vous imposez aujourd’hui vos choix sans débat et sans vote du Parlement. Ce changement de politique publique aura des conséquences graves sur l’ensemble du marché. La parole est à Mme Annick Jacquemet,

Face à la transition écologique, nécessaire, mais parfois brutale, F2J Japy rencontre de grandes difficultés pour se diversifier. En particulier, l’arrêt programmé de la vente des véhicules à moteur thermique d’ici à 2035

exige notamment des investissements significatifs dans la formation pour adapter les compétences des salariés aux nouvelles exigences du marché.

Madame la ministre, quelles mesures concrètes peuvent être prises au plus vite afin d’accompagner financièrement et stratégiquement la diversification de F2J Japy tout en préservant son outil industriel et les emplois locaux ? La parole est à Mme la ministre.

située, vous l’avez dit, à Valentigney dans le Doubs. Cette société spécialisée dans la fabrication de produits métalliques destinés à de grands groupes industriels, en particulier automobiles, compte 102 salariés à ce jour.

En février dernier, la direction de Valeo a brutalement annoncé la cessation anticipée de l’activité du site sarthois d’ici au 25 avril prochain. Quelque 250 salariés sont concernés et attendent les conditions de leur licenciement ou de leur reclassement, sans compter les prestataires affectés par cette fermeture. Dans un bassin de vie comme celui de la communauté de communes du Val de Sarthe, cela signifie qu’aucune famille ne sera épargnée. L’intersyndicale de l’entreprise de la Suze déplore un mépris inacceptable. L’annonce d’une potentielle fermeture a été faite mi juillet, à l’aube des congés, sans égard pour des salariés cumulant en moyenne vingt cinq ans d’ancienneté.

misé. S’y ajoutent des difficultés conjoncturelles, notamment une baisse des volumes et la réorientation des stratégies d’achat des constructeurs vers des pays à plus bas coût. Face à cette chute de son chiffre d’affaires, Valeo a engagé une procédure de recherche de repreneurs pour deux sites.

très attentifs à la qualité du dialogue social, au respect des exigences du code du travail et à la fiabilité des mesures de reclassement qui sont proposées. Plus largement, l’État veille à ce que Valeo maintienne une ambition forte en France.

affichage est pourtant imposé aux fournisseurs d’énergie pétrolière par les arrêtés du 8 juillet 1988 et du 12 décembre 2006. Cette difficulté a déjà été soulevée le 6 juillet 2023 par mon collègue Christian Bilhac, sénateur de l’Hérault, dans une question écrite adressée à M. Gérald Darmanin, alors ministre de l’intérieur et des outre mer. La question étant devenue caduque, aucune réponse n’a été apportée, alors qu’elle soulève un enjeu de régulation essentiel dans un contexte de transition énergétique et de forte croissance du parc de véhicules électriques. Les fournisseurs de recharge pour véhicules électriques appliquent des tarifs fort variables et souvent très élevés en comparaison du coût réel de l’énergie électrique. En effet,

jusqu’à 69 centimes d’euros par kilowattheure sur certaines infrastructures. Ces écarts tarifaires soulignent l’absence de régulation homogène du secteur. Selon l’Autorité de la concurrence, une telle opacité tarifaire empêche les automobilistes de comparer efficacement les offres, au mépris des principes de transparence économique et de protection des consommateurs.

et de garantir enfin la transparence des prix, le Gouvernement envisage t il d’étendre les obligations réglementaires d’affichage des tarifs pour la recharge des véhicules électriques ? La parole

le prix de la recharge électrique dépend de la quantité d’électricité fournie, mais aussi de la puissance de la charge et de la durée de stationnement et d’occupation de la borne. Pour ajouter encore de la complexité, d’autres facteurs, tels que le nombre de véhicules qui se rechargent en même temps, le niveau de charge initiale du véhicule ou encore le modèle de la batterie, ont des répercussions sur la durée de recharge et donc sur le prix.

de ces nouvelles règles, les points de recharge doivent désormais indiquer très clairement le prix de l’énergie par kilowattheure, le prix de la durée d’occupation en minutes et le prix de la session de recharge. À partir du mois d’août, pour les bornes de recharge rapide d’une puissance supérieure à 50

sociale et solidaire. Madame la ministre, je souhaite attirer l’attention du Gouvernement sur des phénomènes de distorsion de concurrence sur le marché du funéraire qui sont liés notamment à l’offensive menée par des opérateurs proposant des contrats obsèques en capital ou des formules de financement d’obsèques à l’avance.

Pourtant, il est constaté que de nombreux organismes financiers influencent les souscripteurs et les familles en deuil dans le choix de leur opérateur funéraire, en les orientant vers des entreprises partenaires, qu’ils rendent seules bénéficiaires, de fait, du tiers payant. Ces partenaires exclusifs sont le plus fréquemment des groupes funéraires. funéraires. Dès lors, les petites et moyennes entreprises, qui représentent pourtant 60 % du marché et plus de 26 000 emplois, se retrouvent exclues. Par ailleurs, certains organismes retardent volontairement le versement du capital prévu lorsque l’opérateur funéraire choisi

Je voudrais, madame la ministre, vous interroger sur ce qui pourrait apparaître comme une déconcertante immobilité politique. J’aurai deux questions. Voilà plus de deux ans, l’un de vos prédécesseurs a annoncé qu’il avait saisi la DGCCRF afin d’enquêter sur les dérives de la, en particulier sur Shein, en matière de sécurité des produits et de loyauté des pratiques commerciales. Ses conclusions, qui étaient attendues pour l’automne 2023, n’ont toujours pas été rendues. Cette situation est d’autant plus étonnante qu’elle contraste avec l’efficacité des actions qui ont été menées par votre ministère à l’encontre de la plateforme en ligne Wish, qui a été déréférencée sur la base de l’article L. 521 3 1 du code de la consommation.